d'effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages pratiques en cabinet d'orthoptie de ville, afin qu'ils puissent connaître la particularité du travail en exercice libéral. seuls les orthoptistes salariés peuvent aujourd'hui recevoir des stagiaires, réduisant de fait la visibilité et l'attractivité de l'exercice libéral auprès des jeunes générations, qui n'ont pas l'occasion de s'y familiariser. Il est donc proposé de lever l'interdiction faite aux libéraux d'accroître leur activité rémunérée, grâce à la présence d'un stagiaire, qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches.

Gouvernement ? S'il est tout à fait légitime d'élargir et de diversifier les offres de lieux de stage pour tous les professionnels, la nature de la relation entre un stagiaire et le professionnel serait tout à fait dénaturée par une telle possibilité

qu'elles aient été commises dans l'enfance ou plus tard, impactent la santé des victimes et sont à l'origine de nombreuses pathologies- souffrances, dépressions, troubles psychiques ou physiques

déjà la remise, chaque année, d'un rapport sur la politique de lutte contre les violences sexuelles. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes comporte une commission « Violences de genre », qui attire l'attention des pouvoirs publics sur des problématiques

utile pour prévenir les grossesses. On le voit, les choses évoluent. Le préservatif va pouvoir être remboursé sur prescription médicale, pour certaines femmes ou certains hommes,

Il est évident qu'un hôpital ne peut pas fonctionner sans anesthésiste. Les chirurgiens ne peuvent alors pas travailler. Quand on manque d'anesthésistes, on est prêt à payer extrêmement cher pour en recruter.

le plafond proposé, fixé à 36,70 euros par mois, serait variable en fonction de l'âge du bénéficiaire, ce qui pourrait être vu comme une rupture à la règle de la sécurité sociale selon laquelle on contribue selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Je souhaitais apporter ces quelques précisions en complément de l'intervention de mon collègue, car nous avions déposé un amendement qui visait à garantir une complète rétroactivité des droits ainsi qu'une continuité de la prise en charge des frais des bénéficiaires des aides à la CMU-C, mais, malheureusement, celui-ci a été déclaré irrecevable.

Madame la ministre, j'imagine que vous allez me répondre que ne pas faire varier le montant de la cotisation en fonction de l'âge pénaliserait les jeunes, qui verraient leurs cotisations augmenter et seraient moins nombreux à recourir au dispositif. Mais le présent

en fonction de leur âge, conformément à une logique assurantielle. Vous proposez de supprimer le critère d'âge pour le calcul de la participation financière.

opté pour un dispositif qui conserve la logique assurantielle de la complémentaire santé, d'où ce critère d'âge, tout en essayant d'en diminuer au maximum les effets sur le coût de la CMU contributive.

améliore l'accès à tous les dispositifs d'aide à la perte d'autonomie, notamment au fauteuil roulant. Pour les personnes handicapées, la couverture sera ainsi de meilleure qualité.

pardonnerez l'expression -de limiter quelque peu les dégâts pour les personnes les plus précaires et d'améliorer une situation difficile.

Les mineurs et les jeunes majeurs qui sortent du dispositif de l'aide sociale à l'enfance sont une population fragilisée, notamment sur le plan de la santé. C'est pourquoi nous avions déposé un amendement qui, nous le regrettons, a été retoqué sur le fondement de l'article 40 de la Constitution. de permettre aux personnes qui sortent du dispositif de l'ASE de bénéficier de la protection complémentaire dès lors qu'elles ne sont rattachées à aucun autre régime d'affiliation à l'assurance maladie jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire. Je pense notamment à celles dont les parents ont été déchus de leur autorité parentale En clair, il n'existe aujourd'hui aucun maintien systématique de l'affiliation à la CMU-C pour ces mineurs et ces jeunes majeurs. Cela engendre des ruptures d'accès aux soins pour cette population particulièrement fragilisée et parfois en voie de marginalisation sociale et familiale.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent article prévoit pour Mayotte une prise en charge intégrale, par l'assurance maladie, du ticket modérateur sur les soins de ville pour les personnes ayant des ressources modestes. Comme vous le savez, 84 % de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. Je voterai bien sûr cet article, mais je souhaite faire quelques observations. Si cette mesure permet de lever tous les frais financiers afférents à l'accès aux soins de ville, encore faut-il que ces soins existent. Or, à Mayotte, ils sont embryonnaires. L'île ne compte, en libéral, que vingt et un médecins, quinze sages-femmes et cinq dentistes, pour une population équivalente à celle de Bordeaux. Nombre d'entre eux sont débordés de travail et épuisés. Il s'agit en fait de désengorger le centre hospitalier de Mamoudzou. Or je crains que les assurés n'aient le sentiment qu'il s'agit de les éloigner davantage encore d'un hôpital en manque de praticiens et surchargé en raison de l'afflux massif d'immigrés illégaux, notamment de femmes venant accoucher. C'est un sujet très sensible à Mayotte. Aussi faut-il rassurer la population. Une nouvelle politique de consultation vient d'être mise en place avec le renforcement des soins sur rendez-vous, la mise en place d'un forfait de dix euros et d'une facture pour les non-assurés sociaux, tout en maintenant la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants. Il faut une politique volontariste de développement de l'offre, tant en ville qu'à l'hôpital. Le Gouvernement a décidé de créer à Mayotte une agence régionale de santé. C'est une avancée majeure. Des travaux d'extension et de modernisation du centre hospitalier sont prévus. La prévention au plus près des populations est indispensable, et je salue la création à Mayotte d'un diplôme universitaire d'animateur en santé communautaire. Quant aux médecins libéraux et hospitaliers, il faut faciliter leur venue et leur maintien dans l'île. Madame la ministre, il se dit que vous préparez un décret en ce sens pour les hospitaliers. Pouvez-vous nous le confirmer ? ? Nous n'attirerons pas les praticiens s'ils craignent pour leur sécurité et celle de leur famille, ni si leurs enfants ne peuvent y suivre une scolarité normale,

Mme Cathy Apourceau-Poly. Malgré la signature de 15 000 contrats d'engagement de maîtrise de leurs tarifs par les médecins en secteur 2, les dépassements d'honoraires médicaux représentent 14 % de l'ensemble des honoraires médicaux, soit près de 3 milliards d'euros annuels. Dans son dernier rapport sur l'avenir de l'assurance maladie, la Cour des comptes juge que les résultats du contrat d'accès aux soins et des options de pratique tarifaire maîtrisée sont « modestes et ambigus », et que l'inflexion observée depuis 2013 est à la fois limitée et coûteuse pour l'assurance maladie. Les dépassements d'honoraires sont un des facteurs principaux de renoncement aux soins pour des raisons financières, ce qui concerne un quart des citoyennes et des citoyens de notre pays. Les spécialistes sont principalement concernés, la moitié d'entre eux pratiquant des dépassements, mais le sont également les établissements de santé à but lucratif, où le taux de dépassement moyen atteint 66 %. Même si cela reste modeste, de médecins hospitaliers publics pratiquant des dépassements, parfois très importants, dans le cadre de leur activité libérale est en nette augmentation depuis dix ans. Nous proposons en conséquence de remplacer la notion subjective de « tact et mesure » par la fixation d'un

Le taux de dépassement est en baisse pour les médecins spécialistes de secteur 2 : 55,4 % en 2011, contre 49,5 % en 2017. Pour la seule année 2017, le taux moyen des dépassements a diminué de 1,6 point. Une dynamique positive s'est donc engagée.

? Il existe déjà des sanctions pécuniaires contre les professionnels de santé. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire est par ailleurs compétente pour connaître des fautes ou abus à l'occasion des soins dispensés aux assurés. Il n'a pas paru opportun

applique le code de déontologie et les sanctions qu'il

chez les jeunes, en répartissant davantage dans le temps les vingt consultations actuellement réalisées avant l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Notre groupe considère qu'il va dans le bon sens, une meilleure politique de prévention de la santé tout au long de l'enfance. Lors de la discussion générale de ce PLFSS, j'ai notamment abordé le sujet de la « précarité menstruelle », à savoir le trop lourd coût que représentent les protections hygiéniques dans le budget des femmes les plus vulnérables. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur un second axe de prévention, l'endométriose, une maladie chronique qui touche une femme sur dix. Cette pathologie,

représente un enjeu sanitaire et d'égalité. C'est un enjeu sanitaire, tout d'abord, lorsque l'on sait les risques pour la fertilité que cette pathologie représente pour les femmes concernées, en plus des souffrances insupportables qu'elle engendre. C'est un enjeu d'égalité, ensuite, lorsque l'on considère l'impact de l'endométriose sur la scolarité des adolescentes qui en souffrent. On l'observe au travers de l'absentéisme scolaire accru que cette maladie cause chez les jeunes filles, portant ainsi atteinte à l'égalité des chances de réussite, en comparaison avec les élèves ne souffrant pas de cet invisible handicap. Pour rappel, en 2016, le ministère de l'éducation nationale signait une convention avec des associations de patientes pour sensibiliser élèves, infirmiers scolaires et enseignants des collèges et lycées. Depuis les campagnes de sensibilisation, l'actuel gouvernement a engagé

Il prévoit que trois des vingt examens aujourd'hui effectués avant les 6 ans de l'enfant soient réalisés entre l'âge de 6 ans et celui de 18 ans, en modifiant l'article L. 2132-2 du code de la santé publique. Dans un avis du 25 mai 2016, le Haut Conseil de la santé publique a considéré que tous les examens au sens de cet article ne sont pas nécessairement médicaux. Ainsi, selon le Haut Conseil, au troisième et cinquième mois, la consultation pourrait être faite par une infirmière puéricultrice diplômée d'État, permettant ainsi de mobiliser des compétences complémentaires à celles des médecins dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, et ce dans un contexte de désertification médicale. Le présent Le présent amendement vise donc à ce que l'arrêté prévu fixe également les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser les différents examens prévus par la loi.

Que répondez-vous aux acteurs de la lutte contre le tabagisme, qui craignent légitimement pour leurs financements ? Enfin, pouvez-vous nous confirmer que l'alcool, deuxième

psychoactives. Précisons tout d'abord que ce plan d'action contre les addictions n'a toujours pas été présenté par le Gouvernement. Il devait l'être en mars, puis en juin dernier, puis il y a quelques semaines,

de cet amendement a un lien direct avec l'intervention, à l'instant, de notre collègue Bernard Jomier. La dilution du fonds actuel de lutte contre le tabac, « chargé de la participation au financement des actions de lutte contre le tabac », dans un fonds dédié à la lutte contre toutes les addictions ne tient aucun compte de la réalité du terrain. Les acteurs de la prévention du tabagisme, pourtant membres depuis l'origine du comité de pilotage du programme national de lutte contre le tabac, ont été exclus de tous les échanges sur la mise en place de ce fonds de lutte contre les addictions. Dévier la lutte contre le tabagisme vers la lutte contre l'ensemble des addictions, sans financement à la mesure des enjeux, affaiblit dangereusement les actions de prévention du plan national de lutte contre le tabagisme 2018-2022 et supprime son caractère prioritaire. Les réponses apportées aux comportements à risque doivent être propres à chaque substance. Si la réduction du tabagisme et de la consommation d'alcool est liée aux politiques visant à encadrer l'offre de ces produits, les drogues illicites relèvent du domaine du soin et de la prise en charge des patients, leur offre étant illégale. la disposition prévue par l'article 38 va entraîner un effondrement du financement des actions de lutte contre le tabac par dilution des ressources. C'est pourquoi il convient de poursuivre un financement efficace de la lutte contre le tabagisme, à la hauteur de ce défi de santé publique. Tel est l'objet du présent amendement.

L'idée d'un fonds élargi ne nous semble pas devoir

veux aussi vous rassurer sur un autre point : ce fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives s'accompagne d'autres fonds dédiés à la prévention des addictions. En 2017, les ARS ont consacré

les autres centres dédiés à la lutte contre les addictions à hauteur de 411 millions d'euros, avec 1,9 million d'euros supplémentaires

qu'il comprend six grands axes de travail : protéger les plus jeunes, mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société, améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic, renforcer les connaissances sur ces sujets et favoriser leur diffusion,

Mme la ministre. L'engagement du Gouvernement d'agir avec détermination dans la lutte contre les addictions outre-mer s'est matérialisé à l'Assemblée nationale par la création d'une section spécifique au sein du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Par cohérence, le Gouvernement souhaite préciser que les actions de la section outre-mer du fonds seront spécifiquement mentionnées dans l'arrêté annuel fixant la liste des bénéficiaires et la destination des sommes versées au titre du fonds. Nous

Cette disposition est entrée en vigueur le 1 juillet 2018. On peut saluer l'impact relatif d'une telle modulation, mais certains industriels

objet de fixer un objectif en termes de pourcentage, afin de rendre la taxe soda pleinement effective et de mieux prévenir les risques que fait peser la consommation de sodas et autres boissons sucrées.

plus la quantité de sucre par hectolitre est importante, plus la taxe est coûteuse. Notre collègue veut changer ce mode de calcul pour taxer le prix de vente, et non plus la quantité de sucre présente dans la boisson, afin de prévenir les stratégies de contournement qui tendent à diminuer la contenance pour limiter le coût de la taxe, tout en maintenant ou en augmentant le prix. Toutefois, ce mode de calcul aurait pour effet de traiter indifféremment,

explication de vote.

Mme Deromedi, concerne le suivi des cancers pédiatriques. Le suivi simple des enfants ayant été traités pour cancer s'étale sur cinq à sept ans. Ensuite, la prise en charge à 100 % est en principe supprimée, sauf en cas de cancer persistant ou recommençant. Par ailleurs, les conséquences des traitements d'un cancer pédiatrique surviennent tardivement ou ne peuvent être détectées qu'après un certain nombre d'années. Par exemple, les séquelles les plus fréquentes n'apparaissent qu'après la puberté. Autre exemple, la stérilité. Ces deux types de séquelles ne sont généralement pas repérés lors de consultations de suivi simple, car les enfants sont trop petits et les séquelles ne sont pas encore développées. De plus, ces jeunes adultes doivent s'approprier leur parcours médical pour se prendre en charge et connaître leurs risques. Il est important de vérifier les procédures de suivi actuellement mises en oeuvre. Cela contribuerait en effet à éviter certaines maladies : pathologies cardiaques ou cérébro-vasculaires, un second cancer, un handicap s'aggravant avec l'âge, etc. Parmi les solutions possibles, on pourrait, par exemple, proposer le bénéfice d'une consultation gratuite

: La parole est à Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à autoriser les pharmaciens à dispenser certains vaccins à prescription médicale obligatoire, dont la liste est fixée par arrêté. En effet, le statut de nombreux vaccins évolue, la prescription médicale passant de facultative à obligatoire. Les pharmaciens d'officine pourraient ainsi participer à la politique de renforcement de la couverture vaccinale et faciliter le parcours de soins des patients.

effet, les dispositions de l'article 39 pourraient rester lettre morte en raison de textes européens prévoyant le passage de l'ensemble des médicaments injectables sous le régime de la prescription médicale obligatoire.

mis en place par les autorités sanitaires sur les vaccins. L'évolution progressive du statut de délivrance des vaccins provient en effet d'une mise en cohérence de la réglementation à l'échelle

et le dépistage des cancers féminins. Par cet amendement, je vous propose de mettre en place une consultation autour de l'âge de 12-14 ans, aussi bien pour les filles que pour les garçons.

! Les actions visant à sensibiliser les jeunes aux infections sexuellement transmissibles et à la vaccination, notamment contre le papillomavirus, peuvent intervenir dans le cadre des cours d'éducation sexuelle ou à l'occasion de la consultation pour les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans sur la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. En outre,

personnaliser les dépistages en fonction des niveaux de risques, notamment pour le cancer du sein et du col, et donc de permettre un dépistage précoce pour les femmes à haut risque.

le suivi des jeunes, en redéployant de 0 à 18 ans les examens de santé obligatoires. Nous venons ainsi de fixer ensemble trois nouvelles consultations : à 8-9 ans, 11-13 ans et 15-16 ans.

Le Gardasil et le Cervarix, recommandés en prévention du cancer du col de l'utérus, « n'entraînent pas de risque accru de maladies auto-immunes », selon une étude de l'assurance maladie.

mettre sur pied une équipe totalement indépendante, qui pourrait d'une façon scientifique mener une expertise sur la toxicité ou pas de ces adjuvants. Il faudrait aussi laisser le choix

du Gouvernement ? Madame Cohen, j'ai beaucoup de respect pour votre travail. Vous travaillez beaucoup, mais, là, je note une incohérence absolument incroyable par rapport au positionnement de votre groupe.

identifié comme première mesure pour éradiquer un cancer que nous pouvons prévenir à 100 % la vaccination HPV chez les jeunes femmes, notamment dans les territoires les plus défavorisés. C'est l'association vaccination et dépistage qui permettra d'éradiquer définitivement un cancer dont on ne devrait pas mourir et dont meurent, particulièrement, je le répète, les populations les plus défavorisées. Madame Cohen, je ne comprends pas votre attitude, qui est de nature à faire peur, alors que, au contraire, vous devriez défendre l'accès à la vaccination pour toutes ces femmes. contribuez aux inégalités de santé en tenant de tels propos, qui ne sont pas raisonnables sur le plan scientifique. Je rappelle que le vaccin contre le papillomavirus a fait l'objet de multiples études à travers le monde. La dernière, la plus belle, est celle qu'a réalisée l'assurance maladie, Santé publique France et l'ANSM,

Cette étude ne montre aucune différence en termes de maladies auto-immunes sauf, pour être totalement précise, quatre cas de maladie de Guillain-Barré en plus dans la cohorte des femmes vaccinées, mais nous savons de longue date que les vaccins, comme les virus, peuvent donner des maladies de Guillain-Barré. C'est un risque connu, qui figure sur le RCP, le résumé des caractéristiques du produit, et qui est de l'ordre de un pour un million pour la plupart des vaccins. Je note d'ailleurs que le vaccin contre la grippe peut donner des Guillain-Barré, mais la grippe elle-même entraîne beaucoup plus de Guillain-Barré que la vaccination. Tout cela est parfaitement connu, parfaitement codifié, scientifiquement démontré. Je le répète, il n'y a aucune maladie auto-immune après la vaccination contre le papillomavirus, en dehors du Guillain-Barré, qui est connu et figure dans le RCP. Je pense donc qu'il faut en finir avec ces mauvais débats. En l'occurrence, madame Cohen, je trouve que votre positionnement est totalement contraire au principe, que vous défendez, d'égalité devant la santé. Bravo ! La parole est à M. Michel Amiel, pour explication de vote.

une façon élégante de contourner cette difficulté, c'est le vaccin. Celui-ci ne protège pas à 100 %, vous le savez. Il y a notamment la myofasciite à macrophages, que vous avez citée,

très souvent, et c'est fort honorable, l'intérêt collectif et l'intérêt général face aux dérives de l'individualisme. Or, sur ce débat de la vaccination, il est justement question de savoir si

conduire à faire primer l'intérêt général sur la liberté individuelle de chacun.

dans ceux qu'ils prennent. De même, pour les vaccins, après la baisse de 2016 à 69 % de confiance, le niveau progresse de nouveau cette année à 71 %, dont 22 % de « tout à fait confiance Le rapport bénéfices-risques associé aux vaccins rebondit également : 52 % des Français considèrent désormais que les vaccins présentent plus de bénéfices que de risques pour la santé. À mon sens, ce taux reste

Notre amendement vise à préciser la nature et le champ des actions qui pourront être mises en oeuvre dans le cadre de l'expérimentation. Nous mettons notamment en avant l'indispensable partenariat avec les acteurs de la santé scolaire. Il s'agira ainsi de financer des actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d'information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l'éducation nationale et les services de santé scolaire. Dans l'article tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, deux régions sont déjà retenues pour l'expérimentation : Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Il a semblé à votre commission qu'il était préférable de laisser à l'État le soin de sélectionner les deux régions pilotes

téléorthophonie, dans le but d'accélérer le déploiement des nouveaux usages de la téléorthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales. Cette expérimentation rechercherait un triple objectif : faciliter l'accès aux soins, notamment dans les zones de désertification médicale ; optimiser le parcours de santé, principalement des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ; renforcer l'efficacité de la prise en charge des patients. Cette expérimentation porterait sur le déploiement de la téléorthophonie pour les patients pris en charge en ville, au sein des établissements hospitaliers et dans des structures médico-sociales, sur plusieurs régions pilotes, pour une durée de trois ans. Elle serait fondée sur un cahier des charges national défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Son pilotage reposerait fortement sur les agences régionales de santé. Elle pourrait notamment s'appliquer au suivi des séquelles des AVC ou dans le cadre de traitement en cancérologie ayant un impact majeur au niveau de la communication du langage et des fonctions oro-faciales, par exemple.

d'engager entre les partenaires conventionnels une réflexion sur la possibilité pour l'orthophoniste d'intervenir à distance auprès des patients la téléorthophonie, d'abord dans le cadre d'expérimentations.

? Nous venons de faire entrer dans le droit commun la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, mais la question de l'accès des auxiliaires médicaux à médicaux à ces pratiques n'est absolument pas cadré. C'est une problématique sur laquelle nous souhaitons travailler, parce que nous avons des demandes multiples : les orthophonistes, mais d'autres professionnels veulent aussi s'inscrire dans cette dynamique.

de la rééducation du langage. Cette profession est très spécifique et demande un lien très fort pour voir des progrès avec les patients. Il y a, certes, une part technique, mais également une

pour rendre obligatoire la vaccination contre la grippe du personnel, en général, exerçant dans des établissements de santé publics, privés, mais également en libéral. Il a été montré, et la Cour des comptes l'a rappelé,

n° 342, le code de la santé publique prévoit déjà que toute personne travaillant dans un établissement accueillant des personnes âgées et exerçant une activité l'exposant à une contamination doit être immunisée contre plusieurs maladies, dont l'hépatite B et la grippe. Toutefois, cette obligation vaccinale peut être suspendue par décret. Un décret du 14 octobre 2006 a ainsi suspendu la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la grippe.

Quand un soignant peut transmettre une maladie potentiellement mortelle chez un de ses malades, c'est vraiment un enjeu déontologique. J'ai, cette année, proposé aux sept ordres des professionnels de santé de signer de signer avec moi une charte d'engagement, pour qu'ils incitent tous les professionnels dont ils ont la charge à se faire vacciner, parce que c'est avant tout, je le répète, un problème déontologique. Je veux revenir sur ce décret qui a été abrogé en 2006. L'histoire est liée en fait à un avis du Conseil d'État qui a, sur la base de la proportionnalité du risque et de l'obligation, estimé que, la vaccination antigrippale n'étant pas à 100 % protectrice entraînant un bénéfice individuel assez faible pour celui qui la recevait- un soignant en bonne santé a peu de risques de mourir de la grippe ; si on lui demande de se vacciner, c'est pour protéger les personnes âgées ou les personnes vulnérables -, il n'était

Cela dit, quand on voit les ravages de la grippe aujourd'hui, l'engorgement des urgences tous les ans au mois de décembre, les dégâts et le coût sociétal, je me pose la question de réinterroger le Conseil d'État sur l'obligation vaccinale des soignants. Pour l'instant, j'ai considéré qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour faciliter la vaccination des soignants dans les établissements de santé, dans les EHPAD. Des circulaires ont donc été envoyées à tous les établissements. Nous essayons vraiment de relancer de façon très proactive cette vaccination. Nous avons demandé aux ordres professionnels de s'engager à nos côtés. Si nous voyons que la montée en charge de cette vaccination est insuffisante, je pense que nous pourrons réinterroger le Conseil d'État sur la possibilité de la rendre obligatoire pour protéger nos aînés et les personnes malades. Au bénéfice de ces explications, je vous propose

mes amendements pour marquer le coup, même si j'ai entendu vos arguments. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, sur le même sujet

le public. Il faut bien trouver une limite. Ce qui compte, c'est que l'on réduise la circulation du virus, que l'on s'attaque aux établissements de santé et aux EHPAD. Je le confirme, dans notre esprit, ce sont bien tous les personnels intervenant auprès des personnes âgées dans les EHPAD

j'entends bien la totalité

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 40 est le seul du PLFSS à évoquer l'accompagnement des personnes handicapées. Son dispositif n'en est pas moins particulièrement ambitieux, en ce qu'il propose une prise en charge financière intégrale d'un parcours de bilan et intervention précoce pour les enfants atteints de troubles du neuro-développement J'ai pu constater, madame la ministre, que la mesure, bien qu'animée des meilleures intentions, n'était pas toujours parfaitement comprise des personnes auxquelles elle s'adresse. Améliorer le champ du diagnostic était indispensable, mais le faire sans mentionner celui du repérage ne pouvait que créer quelques incompréhensions, qu'il nous faudra clarifier au cours du débat. Un autre point doit être soulevé. L'article 40 introduit dans la loi la notion de troubles du neuro-développement, dont je dois signaler qu'elle n'est pas encore intégrée à la classification internationale des maladies, la CIM, telle qu'établie par l'Organisation mondiale de la santé. L'incorporation de cette nouvelle catégorie diagnostique n'interviendra qu'en 2022, lorsque la onzième version de la CIM sera officiellement adoptée par l'OMS.

d'assurer la pleine effectivité de cet article 40 et de faire en sorte que ces diagnostics et ces parcours de bilan puissent réellement donner lieu à des accompagnements, j'insiste, madame la ministre, pour qu'une instruction ministérielle soit rédigée à destination des MDPH. Ces dernières doivent en effet intégrer, avant l'adoption de la nouvelle CIM, cette nouvelle catégorie des troubles du neuro-développement.

qui rassemble des familles d'enfants atteints de troubles du spectre autistique, TSA, ou autres. Ces familles se retrouvent souvent seules à devoir courir les cabinets médicaux pour les dépistages, à monter les dossiers auprès des MDPH, à chercher la meilleure solution pour l'accueil de leurs enfants à l'école, en institut à l'étranger. Chez moi, dans le Pas-de-Calais, les parents se rendent en Belgique. Ce qui m'a le plus frappée, c'est l'isolement dans lequel se retrouvent ces familles, notamment les mères, une fois le diagnostic posé. Entièrement occupées à assurer le meilleur pour leurs enfants, elles arrêtent de travailler et se retrouvent complètement démunies. Elles m'ont expliqué combien, peu à peu, elles se désocialisent. En cette matière, le handicap mental est un poids très lourd à porter, puisqu'il réduit l'autonomie de son porteur. Les différentes lois sur le handicap sont insuffisantes et ne tiennent pas compte des spécificités du handicap mental pour les personnes atteintes et leur entourage. Cet article a le mérite d'exister. En plus d'une meilleure prise en charge des parcours, c'est aussi d'accompagnement par les institutions de référence que les parents Le « ping-pong » entre MDPH, rectorat, CAF n'est pas seulement usant, il peut parfois être préjudiciable. Dans la jungle des dossiers à compléter, la moindre erreur peut en effet d'autant qu'il se passe, malheureusement, plusieurs mois avant que les premiers versements à prestations se mettent en place pour ces familles. La parole Féret, sur l'article. Madame la ministre, je prends la parole sur cet article pour vous dire l'inquiétude de nombre de familles, acteurs associatifs et intervenants auprès d'enfants « dys » et TDAH. L'article 40 vise à créer une nouvelle prestation, prise en charge entièrement par l'assurance maladie, à destination des enfants présentant des troubles du neuro-développement. Cette prestation, sous la forme d'un parcours de soins coordonnés, devra être organisée par des structures dites de deuxième ligne médico-sociales ou sanitaires, lesquelles recevront un « forfait de bilan et intervention précoce ». La mesure s'inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022.

un éventuel amalgame et à une confusion particulièrement contre-productifs pour eux. L'appartenance aux TND ne crée pas une homogénéité des besoins et des parcours. En effet, les troubles « dys » et TDAH, en tant que troubles cognitifs spécifiques, nécessitent des explorations pluridisciplinaires, qui sont étrangères à l'approche psychologique ou psychanalytique. Elles interviennent d'ailleurs généralement après l'âge Le risque d'équivoque et de glissement des repérages pour les enfants « dys » et TDAH vers des diagnostics de TSA est énorme, car ces troubles cognitifs spécifiques, quand ils sont mal identifiés, conduisent très fréquemment à les y assimiler. Comment donc ne pas s'inquiéter en constatant que les suivis proposés seront pilotés par des structures et des professionnels largement orientés vers une approche essentiellement psychologique et, surtout, psychanalytique des troubles ? ? Oui, le dépistage des enfants « dys » et TDAH est essentiel. Oui, les familles ont besoin d'une prise en charge des bilans et des suivis de leurs enfants, notamment en neuropsychologie, psychomotricité et ergothérapie. Il me paraît urgent de mettre en place une concertation sur ces sujets et de faire le lien avec ce qui se passe dans nos écoles, les MDPH renvoyant toujours plus d'enfants « dys » et TDAH vers le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, au détriment du plan personnalisé de scolarisation, pourtant le seul dispositif adapté à des enfants présentant un handicap au sens de la loi de 2005. J'avais d'ailleurs interpellé au Sénat le ministre de l'éducation nationale sur ce sujet lors d'un débat, le mois dernier, sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Les « dys » et TDAH représentent 80 % des enfants porteurs de troubles neuro-développementaux. Ils ne sont pas autistes et méritent un projet qui tienne véritablement compte de la réalité et des spécificités de leurs troubles. La parole

qui est d'intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de développement, afin de limiter le surhandicap. Il est en effet primordial que l'enchaînement des actions de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce soit rapide et fluide. Dans nos territoires respectifs, nous connaissons, hélas, les carences du système, la détresse des familles et de leurs enfants un temps précieux perdu en raison d'un manque de formation au repérage ou de la saturation des structures spécialisées dans le diagnostic, mais également des obstacles à la prise en charge par l'assurance maladie. L'amélioration de la prise en charge grâce à une nouvelle prestation prestation est une excellente nouvelle, dont chacun se félicitera et vous félicitera, madame la ministre ; une prestation de parcours coordonné, prise en charge par l'assurance maladie sans reste à charge et visant à accompagner les enfants avant même l'établissement du diagnostic. Elle permettra d'intervenir rapidement, de réduire les délais de diagnostic et de soulager le poids qui pèse sur les familles contraintes de financer le recours à des professionnels non conventionnés. Elle s'accompagnera des moyens renforcés de la stratégie nationale 2018-2022, avec, au total, près de 400 millions d'euros dédiés à l'amélioration de la réponse aux besoins des personnes, soit près du double de l'enveloppe du troisième du troisième plan. Autre vertu, cette réforme, accompagnée de son décret d'application, renforcera la coordination des professionnels impliqués dans tous les

La PMI est essentielle pour le repérage, la prise en charge précoce et, plus largement, pour notre politique de prévention et de lutte contre les inégalités. Ce réseau de professionnels est une ressource précieuse. La réflexion sur l'organisation de notre système de santé en lien avec les problématiques de cohésion sociale et territoriale devrait conduire à inclure très largement les professionnels de santé des PMI dans les réseaux de soins. J'espère que nous aurons la possibilité d'en discuter hors de la « guillotine » de l'irrecevabilité financière, qui a eu raison de nos amendements « PMI

porté par l'article 40, qui crée un parcours de soins intégré et financé par l'assurance maladie pour les enfants atteints de troubles du neuro-développement. Cette mesure utile risque néanmoins de ne trouver qu'une effectivité limitée si l'étape préalable- et cruciale -du repérage de ces troubles ne fait l'objet d'aucune réforme. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à faire explicitement mention des recommandations de bonne pratique produites par la HAS en février 2018, qui offrent un outil didactique aux médecins de la PMI et aux pédiatres pour leur permettre de détecter ces troubles le plus tôt possible. Quel est l'avis du Gouvernement

Aujourd'hui, tous les troubles du neuro-développement seront bel et bien concernés par cette mesure, mais on tiendra compte de la spécificité de chaque trouble pour l'accès à tel ou tel praticien.

pathologie à la MDPH. On peut tenir les MDPH informées, elles seront forcément destinataires, à un moment donné, du dossier de l'enfant quand le diagnostic sera posé. Nous parlons là d'un repérage et d'une prise en charge précoces avant même la pose du diagnostic et la demande de

est vraiment le point de départ qui nécessite, ensuite, en pluridisciplinarité, le travail sur la globalité de l'enfant porteur de handicap ou de dysfonctionnements.

Cette nouvelle catégorie de troubles, qui ne sera opérationnelle qu'à partir de 2022, englobe de nombreux syndromes, dont les troubles du spectre autistique, les troubles de la déficience intellectuelle et les troubles de l'apprentissage. L'âge de repérage de ces troubles peut fortement varier et n'intervenir qu'au moment de la première scolarité. Or l'étude d'impact de l'article 40 semble insister sur les enfants de moins de 6 ans, alors que de nombreux troubles du neuro-développement ne sont repérés pour la première fois qu'après qu'après cet âge. Par cet amendement, nous entendons sécuriser leur inclusion.

immédiate du moindre symptôme qui oriente vers un centre de niveau 2. Je ne suis pas favorable à une extension

Dans cet article 40, sont uniquement décrits les niveaux 2 ou 3, en omettant complètement les niveaux 1 et 2 en secteur ambulatoire, assurés par des équipes de soins primaires. Pour ces premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est effectuée par le médecin assurant le suivi habituel de l'enfant. Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agréés par l'ARS. Cela risque, d'une part, d'engorger les structures réservées par la Haute Autorité de santé au niveau 3, donc, aux cas très complexes, d'autre part, de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé par le patient. L'article est en contradiction avec les parcours décrits par la Haute Autorité de santé et les recommandations professionnelles. Par cet amendement, nous proposons donc des modifications visant à mettre en conformité l'article 40 avec les recommandations professionnelles définies par la Haute Autorité

Cet amendement vise à rendre obligatoire la conclusion d'un contrat entre les professionnels de santé libéraux et la structure chargée de la coordination du parcours de bilan de l'enfant atteint d'un trouble du neuro-développement ou de problèmes d'autisme. Ce contrat prévoyant notamment un engagement de bonnes pratiques professionnelles, sa signature est indispensable, alors que la rédaction actuelle de l'article 40 se contente de la rendre facultative.

Si j'en crois l'exposé des motifs de l'amendement n° 190 rectifié, il me paraît fondé sur une inquiétude légitime : l'absence de prise en compte des trois stades de prise en charge des troubles du neuro-développement : le repérage, le diagnostic et l'accompagnement. Il est tout à fait vrai que l'article 40 ne concerne que le deuxième et le troisième niveau sans faire mention de l'étape, pourtant essentielle, du repérage. Pour autant, cette absence se justifie en raison de la nature particulière du mécanisme introduit par l'article 40. Le repérage souffre moins d'un défaut de prise en charge financière, puisqu'il est majoritairement effectué par les professionnels médicaux ou sociaux de la petite enfance, que d'un défaut de formation adaptée au dépistage précoce.

variable selon les troubles et peut relever, entre autres, des centres de référence, des centres de ressources, des services de CHU. De même, les définitions scientifiques relatives relatives à ce troisième niveau dépendent du type de troubles : un trouble autistique ou un trouble « dys », par exemple, ne font pas intervenir les mêmes structures. Il ne m'apparaît donc pas pertinent de figer cette organisation dans la loi. ensuite, proposé de revoir la liste des professionnels qui peuvent participer à ce parcours. Sur ce point, je souhaite préciser que le dispositif est ouvert et englobe la totalité des professionnels libéraux impliqués, qu'il s'agisse de professionnels de santé ou de psychologues, qu'ils appartiennent à une profession de santé libérale conventionnée ou non avec l'assurance maladie, maladie, comme c'est le cas des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Il s'agit non de restreindre la pratique libérale actuelle des médecins ou d'autres professionnels, mais, au contraire, d'offrir une prise en charge complémentaire pour les interventions de certains professionnels dont l'exercice libéral n'est pas couvert par l'assurance maladie. enfin, proposé que la prescription porte sur les bilans et interventions, et non sur le parcours. Une telle disposition est vraiment contraire à la façon dont nous envisageons de prendre en charge ces enfants. Le point innovant du dispositif, c'est justement qu'il évoque un parcours global, cohérent

aux familles, dont l'errance en matière de diagnostic fait l'objet de constats récurrents. Elle serait défavorable à la prise en charge globale de l'enfant, pour lequel nous souhaitons maintenir cette notion de prise en charge d'un parcours

de l'enfant atteint de troubles du neurodéveloppement- les CAMSP et les CMPP notamment -, ils proposent d'y adjoindre les réseaux de santé, ce que la commission a jugé judicieux. Le cahier des charges élaboré par l'ARS, en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques, a également recueilli notre assentiment. En revanche, la commission se montre plus réservée sur le nouveau partage des tâches proposé dans cet amendement. L'organisation du parcours n'incomberait plus aux structures elles-mêmes, mais directement à l'ARS, ce qui risque de rendre cette nouvelle offre particulièrement

Les psychologues des structures désignées sont des professionnels reconnus, formés et compétents dans le repérage, le diagnostic et la prise en charge coordonnée des troubles du neurodéveloppement. Leur expérience dans ce domaine est quotidienne. À ce titre, il apparaît cohérent que, outre les médecins, les psychologues des structures désignées puissent également déclencher et coordonner les parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neurodéveloppement. Le guide de la Haute Autorité de santé sur la coordination entre le médecin généraliste et les acteurs du soin en santé mentale encourage la mise en place de parcours dont la coordination pourrait être confiée à d'autres professionnels que les seuls médecins, notamment les psychologues. Ces dispositifs innovants, qui décloisonnent les parcours en santé mentale en ne les limitant plus à la seule référence médicale tout en répondant à l'exigence de coordination et de pertinence des soins, méritent d'être soutenus, car ils peuvent faciliter l'accès aux bilans et interventions précoces pour les enfants souffrant de troubles du neurodéveloppement. Quel

Bien que le financement du soin médical en structure médico-sociale soit défini par circulaire ministérielle et obéisse à des règles théoriquement homogènes, les carences de la réglementation relative au versement direct des dotations aux structures engendrent d'importantes disparités. L'attribution aux structures médico-sociales d'une dotation financière limitative, assortie d'une réglementation permettant une interprétation large des missions de l'établissement ou du service, n'encourage pas les structures à assurer une couverture de soins plus étendue que les actes les plus nécessaires et les incite à renvoyer la personne handicapée vers sa caisse d'affiliation pour le remboursement de tout soin complémentaire, notion elle aussi largement interprétée. Avec l'amorce du virage inclusif, il est particulièrement urgent que la réglementation en vigueur détermine clairement la part qui doit être couverte par l'établissement au titre de sa dotation et ce qui doit être remboursé par la CPAM au titre des prestations libérales extérieures. extérieures. Concernant la prise en charge des remboursements, j'ajouterai que la position des CPAM dans les départements peut être différente selon les situations. Certaines familles doivent donc financer elles-mêmes certains soins non dispensés au sein des structures médico-sociales. Quel est l'avis de la

Notre collègue Philippe Mouiller a très justement identifié la carence réglementaire concernant le périmètre couvert par le forfait de soins dont bénéficient les structures médico-sociales financées par les ARS. Cette indétermination est à l'origine de nombreux contentieux entre les établissements et les caisses de sécurité sociale, vers lesquelles les familles se tournent pour le remboursement d'actes non inclus.

En réalité, nous partageons tous l'objectif des auteurs de cet amendement. Nous avons donc d'ores et déjà engagé les travaux entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les services du ministère afin d'harmoniser l'interprétation des dispositions existantes et de faire évoluer la réglementation.

Cet amendement assez technique vise à permettre, à titre expérimental et pour une durée déterminée, un conventionnement entre les différentes autorités tarifaires des structures cofinancées afin d'organiser la délégation de la compétence tarifaire au profit de l'une d'entre elles uniquement, ce qui pourrait s'inscrire notamment dans le cadre du déploiement de la démarche des territoires 100 % inclusifs.

prégnant du cofinancement, que l'on observe autant dans le secteur du grand âge que dans celui du handicap, est l'une des principales causes de la rigidité et de l'inadéquation de l'offre aux besoins qu'elle est censée satisfaire. Cet amendement tend à apporter une première réponse

Or les CMPP comme les SESSAD, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, sont en nombre insuffisant pour faire face à la demande, qui ne cesse de croître et à laquelle nous devons répondre de façon concrète et matérielle. De ce fait, les délais d'attente sont extrêmement longs, souvent supérieurs à un an, et l'épuisement des parents et de l'enfant se ressent cruellement.

Un diagnostic tardif engendre également des dépenses très lourdes pour la société, au travers de l'éducation nationale ou de la sécurité sociale. Pour pallier cette carence de structures surchargées et soulager les inquiétudes des parents, des enfants et des

La prise en charge de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique est assurée à hauteur de 100 % dès lors que le handicap a été reconnu. Toutefois, une situation de handicap psychique est très souvent accompagnée de pathologies associées, telles que l'obésité, le diabète ou des maladies cardiovasculaires. En plus

Les mots, même hâtifs, laissent parfois quelques traces, et je préfère de très loin ceux par lesquels vous m'avez répondu lundi dernier, en indiquant que le Gouvernement entendait sortir l'accompagnement du grand âge d'un carcan médical rarement adapté. souscris d'autant plus volontiers, madame la ministre, qu'étant moi-même médecin, je sais autant mesurer la valeur d'un acte médical que ses limites. Il faut Il faut qu'à cet égard notre unisson soit irréprochable. La réponse médicale jusqu'ici communément apportée au défi du grand âge, fruit d'une myopie qui nous fait encore confondre la vieillesse et la maladie, crée peut-être plus de maux qu'elle n'en guérit. Dépendre n'est pas toujours souffrir

qu'entre eux. Ainsi, d'un département à l'autre, les tarifs et les conditions de prise en charge varient, tandis que la clôture des budgets devient un vrai casse-tête pour les établissements. Ce sont les salariés qui en paient le prix. Ils sont descendus dans la rue pour la première fois ce printemps. Devant la grogne du personnel et des familles, vous avez, madame la ministre, annoncé une neutralisation de la réforme et des concours financiers importants. Certes, mais nous considérons que cette réforme, dans sa matrice même, n'est pas la bonne : il faudrait revoir à la hausse les moyens alloués et, notamment, enfin lancer une politique ambitieuse de l'âge, incluant tous les aspects de la problématique du vieillissement. Par ailleurs, la lumière n'est toujours pas faite sur les conséquences de cette réforme de la tarification. Vous mettez en avant, madame la ministre, que la perte subie, notamment, par les EHPAD publics au titre de la dotation dépendance serait en quelque sorte compensée par l'augmentation du forfait soins et les mesures en faveur du financement de postes d'infirmière de nuit. Mais, le compte n'y étant pas, c'est l'austérité qui s'impose

Même si, l'année dernière, j'ai pu dénoncer en commission des affaires sociales les effets dommageables de la réforme tarifaire au moment de sa première application, le Gouvernement a, depuis lors, dégagé d'importants moyens financiers pour les contrer 116 millions d'euros ont ainsi été consacrés en 2018 au rattrapage financier des établissements publics dont la somme du forfait soins et du forfait dépendance était affectée négativement.